la séance est retransmise en direct sur France 3, Public Sénat, le site internet du Sénat et Facebook. J'appelle chacun de vous, mes chers

tel qu'il figurait en loi de programmation des finances publiques, tout en soulignant la modestie dudit objectif. Surtout, elle nous appelle à la vigilance et à la mobilisation pour l'avenir, soulignant que quatre pays restent en déficit excessif : l'Espagne, le Portugal, la Grèce et la France.

et à l'effort demandé aux collectivités territoriales, avec la réduction des dotations de l'État. Ma question est donc double : comment pouvons-nous faire face à une remontée éventuelle des taux d'intérêt, au moment où le décalage des taux entre la France et l'Allemagne est passé de 27 points à 54 points de base entre les mois de septembre et de décembre ? Y a-t-il des réformes structurelles que vous regrettez de ne pas avoir menées au cours de la législature ?

Vous avez bien rappelé la réduction du déficit public, même si le rythme et l'ampleur peuvent en être commentés de façon diverse.

de la santé. Hier, le Conseil d'État a enjoint au Gouvernement de prendre, dans un délai de six mois, des mesures pour rendre disponibles les vaccins contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite, les trois seuls vaccins obligatoires. Actuellement les laboratoires associent ces trois vaccins à d'autres, si bien que, pour se mettre en conformité avec la loi, il faut recourir à des vaccins hexavalents, qui vaccinent aussi contre la coqueluche, l'et l'hépatite B. Au passage, cela permet aux laboratoires d'augmenter leurs marges. Le Conseil d'État a été on ne peut plus clair et a demandé au Gouvernement de permettre l'application stricte de la loi : trois vaccinations sont obligatoires et pas davantage, même si les autres sont, je le rappelle, très fortement conseillées. termes de cette décision, « la loi, qui n'impose que trois obligations de vaccination, implique nécessairement qu'il soit possible de s'y conformer en usant de vaccins qui ne contiennent que ces trois vaccinations. »

hypothèse du reste évoquée par le Conseil d'État lui-même dans son ordonnance ? Enfin, je tiens à préciser que nous partageons entièrement l'analyse du Conseil d'État, qui a écarté l'argumentation des requérants sur les risques allégués des vaccinations non obligatoires, soulignant « qu'aucun élément sérieux n'est apporté sur l'existence d'un risque d'atteinte à l'intégrité de la personne et de mise en danger d'autrui. » Le Gouvernement a-t-il l'intention de renforcer sa politique vaccinale, tordant ainsi le cou à nombre d'idées reçues et de préjugés qui peuvent mettre en danger la santé de nos concitoyens

est l'un des grands succès de notre politique de santé publique. Il ne faut ni oublier ni banaliser les fléaux qu'elle a permis d'éradiquer. Dès le mois de janvier 2016, Marisol Touraine a annoncé un plan de rénovation de la politique vaccinale destiné à mieux informer les professionnels et le grand public, à améliorer la gouvernance de la politique vaccinale et à sécuriser l'approvisionnement, et ce afin de renforcer la confiance dans la vaccination. Un comité d'orientation indépendant, présidé par le professeur Fischer, a également été chargé d'organiser une grande concertation citoyenne sur la vaccination en s'appuyant sur un jury citoyen et un jury de professionnels de santé, ainsi que sur les experts et acteurs de la vaccination. Après plus de 10 000 contributions en ligne, des recommandations ont été présentées le 30 novembre dernier. Celles-ci font actuellement l'objet d'une expertise juridique et financière

les services du ministère et l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pour que l'État puisse la mettre en oeuvre dans le délai imparti. D'un point de vue pratique, je rappelle qu'il existe déjà un kit disponible gratuitement pour assurer la vaccination avec les seules

en tenant compte des recommandations de la concertation citoyenne, et pourrait à terme faire évoluer le cadre législatif sur lequel s'est fondé le Conseil d'État

jeudi dernier, Théo, 22 ans, jeune homme sans histoire, fils d'une famille honorablement connue, a été gravement blessé lors d'une opération de contrôle à Aulnay-sous-Bois. Il affirme avoir été victime d'insultes racistes, de coups et avoir subi un viol. Hospitalisé, opéré en urgence, il s'est vu prescrire soixante jours d'incapacité totale de travail. Parmi les quatre policiers mis en cause, l'un a été mis en examen pour viol, les trois autres pour violences volontaires en réunion. Les faits reprochés à ces quatre policiers rejaillissent injustement sur tous leurs collègues, hommes et femmes sans reproche, dévoués à leur tâche, toujours plus difficile, en butte eux-mêmes à des attaques parfois extrêmement violentes. Pour le Défenseur des droits, « cette dramatique affaire [ ...] illustre les conflits qui naissent parfois des contrôles d'identité. » Et il continue de réclamer que ces contrôles

il faut reconstruire la confiance brisée entre les habitants de certains quartiers et leur police. Ma question est simple. Monsieur le ministre, ne conviendrait-il pas, sans tarder, de rappeler à chacun ses devoirs, de rompre avec certaines pratiques discriminatoires et de faire prévaloir en toutes circonstances l'État de droit ? ? Ne vous paraît-il pas nécessaire de restaurer une police de proximité dûment formée, soucieuse avant tout de connaître et de protéger les citoyens dont elle a la charge ? La

tout ce qui devait lui être transmis l'a été. Je n'ai pas à juger de la rapidité de l'enquête, mais je souhaite qu'elle puisse aller le plus vite possible pour établir la vérité des faits.

et conduits devant la justice. Je veux un équilibre parfait : il n'y a pas dans nos quartiers, comme partout ailleurs dans notre pays, de place pour ceux qui agressent les symboles de la République que sont les personnes dépositaires de l'autorité, de la même façon qu'il n'y a aucune place pour ceux qui ne respecteraient pas les valeurs de la République dans la façon dont ils exercent la mission et l'autorité que nous leur avons confiées. Sur ce point, je veux

doublement des crédits du ministère de l'intérieur sur la question du rapprochement entre la police et la population et la mise en expérimentation prochaine, quand les policiers en seront dotés, du système de caméra mobile, qui, à mon sens, peut présenter le double avantage d'apaiser les interventions

de votre réponse. La tâche est lourde et le chemin sera long, mais espérons que cet acte d'une extrême violence aidera le Gouvernement à prendre les décisions

Face à cette violence inouïe, qui peut être qualifiée d'acte de barbarie, nos pensées et notre compassion vont bien sûr vers Théo, sa famille et ses proches, qui vivent un moment très douloureux. Aujourd'hui, quatre agents de la brigade spécialisée de terrain, Le Défenseur des droits a ouvert une enquête. Et pour cause : d'après ses déclarations, le jeune homme aurait fait l'objet, en plus des coups et du viol, de moqueries, de crachats et d'injures racistes. Cela est profondément révoltant ! Malheureusement, ces faits ne constituent pas un événement tragique et isolé ils font écho à des pratiques pour le moins douteuses de contrôle policier et d'interpellation bien connues dans les quartiers populaires. Mon propos en l'occurrence n'est pas de remettre en cause le travail et la déontologie de l'ensemble de nos forces de sécurité, dont nous reconnaissons la qui plus est dans le contexte actuel et avec le peu de moyens dont elles disposent. Mais une tension permanente, dont témoignent les forces de l'ordre et les citoyens, existe dans ces quartiers. Nous reconnaissons la dégradation des conditions de travail de la police de terrain, mais il convient aussi d'entendre les voix des nombreuses associations et des citoyens, voire du Défenseur des droits lui-même. Tous évoquent des contrôles d'identité discriminatoires, parfois répétés, voire systématiques. Les palpations de sécurité sont souvent faites hors des règles du code de déontologie des forces de sécurité, et s'apparentent trop fréquemment à une véritable atteinte à la dignité humaine. Monsieur le ministre, certes, il faut rester serein, mais comment ignorer que, lorsque certains sont soumis à la justice expéditive de la comparution immédiate, d'autres bénéficient d'une réelle instruction ? C'est incroyable ! La justice, aussi, doit être la même pour tous ! Il faut revenir aux réalités du terrain et, surtout, remettre à plat la doctrine et les pratiques du maintien de l'ordre en France, avec le retour d'une véritable police de proximité, recrutée et formée pour ces missions. Dans ce cadre, de mettre en place d'urgence le récépissé de contrôle, afin d'en finir avec les contrôles au faciès. Ces mesures sont attendues depuis cinq ans. Pourquoi ne pas utiliser le projet de loi Sécurité publique actuellement en discussion pour les faire adopter ? Oui, il faut rétablir la confiance, afin qu'il n'y ait plus de Théo, d'Alexandre, d'Ahmed Selmouni ou d'Adama Traoré

Avec le Brexit, l'Union est confrontée à la crise la plus grave qu'elle ait eu à connaître depuis sa fondation. Un divorce, après quarante ans de vie commune qui ont tissé des liens très forts, est nécessairement difficile, douloureux, complexe. Pour autant, nous devons être fermes

L'Union doit aussi faire face à des difficultés du côté transatlantique. Pour le locataire de la Maison-Blanche, « cela n'a aucune importance [ ...] que les Européens soient unis ou non ». « Le Brexit va être une chose merveilleuse » d'autres pays vont quitter l'Union européenne », qui est « un instrument au service de l'Allemagne ». Ces déclarations surprenantes, choquantes, montrent que le président des États-Unis nouvellement élu ne maîtrise pas bien la matière européenne.

Pour relever les nombreux défis qui sont devant eux, les États membres de l'Union doivent faire bloc et réaffirmer les valeurs sur lesquelles repose la construction européenne.

souhaite mettre en avant dans la perspective des prochains sommets européens

quand l'un de ses membres les plus importants, à savoir l'Allemagne, est mis en cause par le nouveau président américain. Quand le nouvel ambassadeur désigné par l'administration Trump auprès de l'Union rappelle qu'il a été auparavant en poste auprès de l'Union soviétique et qu'il souhaite que l'Union européenne connaisse le même sort que celle-ci, nous devons d'abord affirmer notre unité. C'est pourquoi

que nous avons accompli de grandes choses ensemble, après tant de guerres qui avaient déchiré le continent, que les valeurs qui ont fondé le projet européen, c'est-à-dire la paix, la coopération, la démocratie, les droits de l'homme, restent actuelles et indispensables pour le continent. Il faudra surtout réaffirmer que nous avons l'ambition

Aujourd'hui, la confiance revient à Calais. Eurotunnel bat des records de traversées pour ce qui concerne les camions. Les Britanniques fréquentent de nouveau les commerces de Calais. Mais- car il y a un « mais -les migrants sont de retour, surtout les mineurs, attirés par la Grande-Bretagne. Qui plus est, à quelques kilomètres de Calais, à Grande-Synthe, 1 500 migrants vivent dans un camp où les passeurs font la loi, nous dit-on. La violence s'y est installée.

Enfin, dernière question, avec le Brexit, la frontière de la Grande-Bretagne étant plus que jamais à Douvres et pas à Calais, ne pensez-vous pas nécessaire de revoir les accords du Touquet ?

de Belfort. Une mobilisation très forte s'est ensuivie. Le 4 octobre, le Gouvernement a annoncé un plan de sauvetage que les élus, dans leur immense majorité, soutiennent fermement. Ce plan contient un volet « nouvelles commandes » sur lequel nous attendons encore des garanties, car rien n'est assuré. Qu'en est-il de la fragilité juridique du dispositif exposé dans une note de Bercy, censée être confidentielle, mais parue lundi dans un grand quotidien national ? Cette note, que M. Sirugue a démentie, a réveillé de mauvais souvenirs chez les salariés d'Alstom et dans la population du Territoire de Belfort. J'ai la conviction que sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, certaines officines, qui ne souhaitent pas voir aboutir cet accord, sont à la manoeuvre, afin de le discréditer. Nous serons toujours extrêmement vigilants sur la bonne réalisation de cet accord et sur le respect de la parole de l'État. Il faut désormais des actes. Les collectivités locales jouent le jeu. Elles avancent et tiennent leurs engagements. Il faut que le 17 février prochain, lors de la réunion du comité de suivi, des engagements forts soient pris par l'État en direction d'Alstom et de ses salariés. Les investissements que doit réaliser Alstom sur le site de Belfort dépendent, bien entendu, de nouvelles commandes, lesquelles, pour l'heure, n'arrivent pas. Je suis d'autant plus inquiet quand je vois que le conseil d'administration de SNCF Mobilités

faire de la mixité sociale un objectif essentiel de la politique éducative, réexaminer la sectorisation en introduisant la notion de choix multi-collèges et moduler les dotations financières

la mission de veiller à la mixité sociale au sein des établissements scolaires. Dès novembre 2015, Mme la ministre a impulsé la mise en oeuvre sur le terrain de cette politique publique essentielle, mais difficile, Cela a été fait de la meilleure façon possible : résolument, mais avec prudence, et sous la forme d'expérimentations, en associant en tout premier lieu les acteurs de terrain. La dernière enquête PISA nous le rappelle, si la France s'affiche au sein de l'OCDE comme le pays où l'origine sociale pèse le plus lourdement sur la réussite des élèves, la ségrégation scolaire y est pour beaucoup. Or la mixité a des effets positifs sur tous les élèves, tant sur les résultats scolaires qu'en matière de cohésion sociale. Mais, nous le savons cette politique publique ambitieuse, si elle n'est pas préparée, expliquée aux parents, accompagnée sur le long terme, provoque des réactions souvent vives. Aujourd'hui, 46 départements ont défini 82 territoires pilotes.

Oui, la ségrégation sociale est en France une réalité ! Et je pense que le sujet vaut la peine que l'on s'y attarde parce que nous en connaissons l'ampleur et la cartographie. Si 10 % des collèges accueillent moins de 15 % d'élèves d'origine sociale défavorisée, 10 % en accueillent plus de 63 %. Cela signifie que des générations d'élèves grandissent dans notre pays et fréquentent la même institution sans jamais véritablement Et nous voyons mal comment l'école pourrait transmettre une appartenance commune à la République sans lutter contre les processus d'exclusion. C'est pourquoi Mme Vallaud-Belkacem a soutenu la question de la mixité sociale scolaire comme l'un des enjeux de la mixité dans nos quartiers populaires. La carte scolaire est l'une des réponses opératoires. Certains voudraient une carte plus rigide, au risque d'entraver la mobilité sociale. D'autres veulent assouplir celle qui existe, alors même que les études ont montré son importance et sa pertinence.

Des solutions adaptées aux territoires ont été élaborées et sont mises en oeuvre à travers la resectorisation des élèves, la mise en place de secteurs multicollèges et l'évolution de la carte des formations. Et cela marche, madame la sénatrice ! La ministre a donc souhaité étendre ce dispositif dans 82 territoires, autour de 248 collèges. Dans les 46 départements concernés- n'en déplaise à certains ! -, l'engagement des élus a été transpartisan. Et je souhaite ici m'associer à Mme Najat Vallaud-Belkacem pour saluer l'implication des élus locaux, tant ce sujet est également important pour la secrétaire d'État chargée de la ville que je suis.

des finances publiques, les seuils réglementaires s'élèvent à 180 000 euros pour les acquisitions hors expropriations contre 175 000 euros auparavant et à 24 000 euros de loyer annuel pour les prises de bail contre 12 000 euros auparavant.

et les autres collectivités locales tenues à consultation des domaines dans ce cadre. S'agissant des communes de moins de 2 000 habitants, elles sont dispensées de consulter le service France Domaine en matière de cession. cession. Je souhaite donc que vous puissiez, monsieur le secrétaire d'État, apporter des précisions aux maires des communes rurales qui viennent d'être informés de ce changement par vos services et qui s'inquiètent des conséquences de cet arrêté. en effet nombreux à faire appel aux domaines et à leurs agents pour obtenir des conseils gratuits et des évaluations incontestables lors d'échanges de terrains, de cessions ou de ventes, même sur des montants

mais est-ce une raison pour que la signature officielle du Comité Paris 2024 affichée sur la tour Eiffel soit « » ?

N'aurions-nous pas pu trouver autre chose, en français, pour résumer l'esprit de notre candidature, dans le pays de Pierre de Coubertin, restaurateur des jeux Olympiques, qui avait tenu à ce que le français en soit la langue officielle ?

dites donc en français que « Paris est une fête », comme l'a jadis écrit- c'est le titre célèbre de l'un de ses livres -Ernest Hemingway. Vous verrez alors que chacun comprendra En renonçant à signer notre candidature dans notre langue, vous proclamez que la France renonce au rôle international du français. Une fois de plus, vous désespérez nos amis québécois et africains qui ont, avec nous, le français en partage et qui en sont fiers, eux Monsieur le secrétaire d'État, qu'allez-vous faire pour corriger cette erreur, qui est même plus qu'une erreur, une faute !

Le Comité international olympique a créé des conditions pour une candidature. Il faut le savoir, la candidature officielle a été déposée voilà plus d'une année. Au cours d'un stade intermédiaire, nous devions déposer un deuxième dossier.

et porte sur le cadre professionnel et les perspectives des métiers d'aide à domicile. Récemment, au mois de décembre 2016, le Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, s'inquiétait des conditions d'intervention des aides à domicile dans mon département, la Somme. Dans un courrier adressé au président du conseil départemental, il s'interrogeait en effet sur les conséquences des décisions du département dans ses modalités de déploiement des aides à domicile en direction des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, l'APA.

un élément nouveau et tout récent est à verser au dossier. En effet, le tribunal d'Amiens, en statuant sur plusieurs dossiers et recours faits par des personnes âgées, vient d'ordonner,

à domicile. En affaiblissant le mode prestataire qui permet de salarier ces intervenants dans des associations ou des services, on précarise fortement une profession déjà très difficile : multiplication des employeurs, diversité des contrats de travail, convention collective différente, organisation du temps de travail morcelée, indemnités de transport ou droit à la formation diminués ... Ces auxiliaires de vie, qui gagnent en moyenne de 800 à 1 000 euros par mois, ont besoin, au contraire, d'accompagnement et de cadre professionnel stable.

des personnes âgées pour faire respecter la loi, respecter les personnes âgées et leur libre choix, sans oublier celles et ceux qui travaillent à leur service, c'est-à-dire les aides à domicile. La loi est passée. Le droit a été dit. Il s'agit maintenant de rendre leur dignité à ces personnes âgées. Monsieur le sénateur, vous avez raison : ce métier d'aide à domicile est un véritable enjeu pour notre pays, car, dans dix ans, un tiers de notre population aura plus de 65 ans. Pour

Elle dresse un bilan très sévère, relevant que la décision de Mme Royal, d'abord de suspendre l'écotaxe, puis de résilier le contrat de partenariat, a été prise- je cite M.

reconnaît-elle devant la représentation nationale le grand gaspillage budgétaire dont elle est responsable dans cette affaire ? Quelles suites entend-elle donner au rapport accablant de la Cour des comptes ?

La séance est reprise. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi relative à la lutte contre l'accaparement des terres agricoles et au développement du biocontrôle est parvenue à un texte commun. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de réunion d'une commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière pénale. En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du mercredi 8 février

l'année 2017 constitue un tournant très important pour l'AFPA, l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes. Depuis 1946, l'AFPA n'a cessé d'agir au service des politiques de l'emploi et de la formation, en

aux qualifications, y compris pour les personnes les plus éloignées de l'emploi et de la formation, quel que soit leur territoire.

le Gouvernement a été convaincu de la nécessité d'accompagner l'AFPA afin qu'elle puisse répondre aux enjeux actuels en s'appuyant sur ses points forts tout en continuant d'assurer un service public au bénéfice de la collectivité nationale.

Le projet du Gouvernement s'appuie sur un constat : pour des raisons tant économiques que juridiques, il est indispensable de faire évoluer en profondeur le statut de l'AFPA qui est, depuis l'origine, une association. Il s'agit tout d'abord de répondre à la déstabilisation du modèle économique de l'AFPA. La compétence des conseils régionaux en matière de formation professionnelle a été progressivement renforcée, avant de devenir exclusive.

une réduction significative de son chiffre d'affaires. À partir de 2009, elle a connu une période très difficile de déséquilibre financier croissant, qui a fini par menacer son existence même. À la fin de la précédente législature, l'AFPA était au bord du défaut de paiement, sans vision stratégique ni espoir de redressement.

comme M. le rapporteur l'a souligné dans son rapport. En effet, au sein de cette structure se conjuguent des activités relevant du domaine concurrentiel et des missions de service public que l'État doit financer et auxquelles le Gouvernement, comme vous-mêmes, attache une importance considérable.

La transformation de l'association en établissement public industriel et commercial, ou EPIC, permet précisément de résoudre cette difficulté en distinguant clairement les missions de service public des activités soumises à la concurrence, qui relèvent des filiales. Une fois posé le constat de l'impossibilité du, le Gouvernement a décidé, pour ne pas laisser péricliter l'AFPA, de s'engager de façon extrêmement ferme, forte et déterminée dans un processus de transformation. Il a accompagné ce processus, depuis 2012, en plusieurs étapes, en ayant toujours le souci de maintenir le potentiel humain technique, le savoir-faire et les valeurs de l'AFPA, et de les mettre au service des politiques de formation dans notre pays. En 2012, le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, sur la proposition de Michel Sapin, alors ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, s'est engagé, pour les raisons stratégiques que je viens d'évoquer, dans ce processus de transformation. Il a affirmé sa volonté de développer un projet pérenne permettant la refondation de l'AFPA. Cette démarche a été confortée par la loi du 17 août 2015, défendue par François Rebsamen, qui a inscrit l'AFPA dans le périmètre du service public de l'emploi, en pleine cohérence avec les objectifs politiques du Gouvernement. loi lui confie des missions de service public et autorise le Gouvernement à engager le processus de transformation de l'association en EPIC. L'ordonnance du 10 novembre 2016, vecteur de cette transformation, constitue l'aboutissement du processus

Le positionnement de l'établissement public au sein du service public de l'emploi repose sur une définition extrêmement claire des missions de service public, financées par l'État à hauteur de 110 millions d'euros en loi de finances initiale pour 2017. Ces missions sont décrites dans deux articles complémentaires de l'ordonnance. Le premier réaffirme la compétence historique de l'AFPA comme acteur de la politique de certification, ainsi que le sens même de son utilité sociale dans la lutte contre les inégalités d'accès à la formation, qu'elles soient sociales, territoriales ou encore liées au genre. Le second article identifie, parmi les missions de service public déjà présentes dans le programme d'activité de service public de l'association, celles dont le développement revêt une importance clé, dans le monde d'aujourd'hui, pour la compétitivité de notre économie et la réponse aux besoins de formation des personnes. Ces besoins

dont vous connaissez l'importance, afin d'accompagner les personnes qui en ont le plus besoin. Les autres activités de l'établissement ne bénéficieront pas de dotations de l'État et s'exerceront dans le cadre de deux filiales : l'une consacrée à la mission de service public concurrentiel de formation des demandeurs d'emploi ; l'autre, à la mission de formation des salariés. Ces filiales relèveront pleinement du droit des sociétés. Les conventions et accords collectifs applicables avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance s'appliqueront à l'ensemble des personnels de l'établissement. Il est en outre prévu de négocier une convention collective permettant la constitution d'une unité économique et sociale dotée d'un comité central d'entreprise commun à l'établissement public et à ses filiales. Outre la définition des missions de l'établissement, l'ordonnance fixe les modalités de gouvernance. Celles-ci respectent le quadripartisme : sont représentés au

le 1 janvier 2017, date d'entrée en vigueur du statut d'établissement public. Enfin, l'ordonnance règle la question du patrimoine immobilier de l'AFPA, qui était posée de longue date, en organisant les conditions du transfert vers l'EPIC, lors de sa création, de biens de l'État utilisés, jusqu'à présent par l'AFPA. Ces dispositifs se sont concrétisés par la dévolution, au 1 janvier 2017, de 116 sites de l'État vers l'EPIC, en conformité avec les exigences posées par la Commission européenne. Cette dévolution permettra à l'EPIC d'assurer une présence sur tout le territoire, comme le nécessite l'exercice de ses missions de service public.

mais aussi à ceux des entreprises, dans le cadre de projets stratégiques définis au cas par cas. L'ordonnance soumise à la ratification du Parlement est donc un texte équilibré, solide et respectueux des compétences des conseils régionaux et des partenaires sociaux.

en vigueur et soit adapté aux exigences d'aujourd'hui. Dans ce cadre ainsi rénové et clarifié, il appartient désormais à la direction de l'établissement et à sa communauté de travail de bâtir un projet de développement régional, site par site, région par région, et à l'échelle nationale.

la voie de la facilité, mais celle d'une ambition stratégique forte, avec des objectifs politiques clairs. Oui ! Les missions de service public du nouvel établissement ont été volontairement et précisément définies, en prenant en compte à la fois les valeurs et les acquis de cet

et sans concession sur un sujet qu'il connaît bien et depuis longtemps. Je veux souligner ici la qualité de son rapport. Je voudrais aussi remercier les membres de la commission des affaires sociales

le texte que nous examinons aujourd'hui devrait clore une longue période d'incertitude sur l'avenir de l'AFPA, principal opérateur de la formation professionnelle en France, qui accompagne les mutations de l'économie de notre pays depuis la Libération. Le présent projet de loi ratifie l'ordonnance du 10 novembre 2016 qui a transformé l'AFPA, au 1 janvier dernier, en établissement public à caractère industriel et commercial. est conforme à l'habilitation que le législateur a conférée au Gouvernement à ce sujet dans la loi Rebsamen du 17 août 2015. Pour autant, cette nouvelle agence reste confrontée aux mêmes difficultés que celles qui avaient conduit l'association au bord de la faillite en 2012. Il est donc urgent de saisir l'opportunité offerte par ce changement statutaire pour réinventer un organisme de formation compétitif sans renier l'utilité sociale qui a fait sa force. Au cours de mes travaux, j'ai eu l'occasion de rencontrer l'ensemble des acteurs clés de ce dossier. J'en ai acquis une conviction unanimement partagée l'inaction aurait à court terme condamné l'AFPA. Au vu du déclin de son activité et de sa situation financière très dégradée, elle n'aurait bientôt plus été en mesure de faire face à ses obligations. Depuis plus de dix ans, l'AFPA est en effet victime d'un double phénomène qui a bouleversé son modèle économique : d'une part, l'entrée dès 2008 des activités de formation dans un champ purement concurrentiel, d'autre part, la décentralisation aux régions des subventions de l'État qui finançaient des formations en faveur des demandeurs d'emploi.

son chiffre d'affaires est passé d'un milliard d'euros à 710 millions d'euros, tandis que le nombre de stagiaires a chuté de 25 %. Cette baisse est encore plus prononcée s'agissant des seuls demandeurs d'emploi : elle est de l'ordre de 35 % sur cette même période. Quant à la part de marché de l'AFPA dans les commandes de formation des conseils régionaux, elle est passée de 42 % en 2010 à 25 % l'an dernier. Le plan de refondation engagé en 2012 a eu des résultats mitigés et n'a pas permis de redresser la situation. S'il témoigne d'une réelle prise de conscience des difficultés structurelles de l'association, il ne les a pas résolues. de l'AFPA ont continué à se creuser, passant de 91 millions d'euros en 2012 à 152 millions d'euros en 2015. Le caractère hybride de l'association,

Respecter la réglementation communautaire en matière d'aides d'État et de services d'intérêt économique général, ou SIEG, tout en assurant le transfert à l'Agence des biens jusqu'à présent mis à la disposition de l'AFPA par l'État tel était l'objectif de l'ordonnance du 10 novembre 2016. Force est de constater qu'elle offre de solides garanties en la matière. La ligne de crête était très étroite, mais le Gouvernement, dans le cadre d'un dialogue approfondi avec la Commission européenne et le Conseil d'État, a su trouver un équilibre satisfaisant entre des attentes parfois divergentes. Les tutelles et la nouvelle direction de l'Agence devront rapidement définir des critères pour calculer les compensations qui lui sont attribuées pour l'exercice de ses missions de service public. Ces dernières ont d'ailleurs été étoffées, dans le prolongement de celles qui sont historiquement attribuées à l'AFPA. Il est essentiel que l'État ne se désengage pas financièrement de son nouvel opérateur le risque serait qu'il ne puisse plus alors assumer l'intégralité de ses missions. À l'inverse, un niveau de subvention trop élevé pourrait être qualifié de surcompensation par la Commission européenne et contraindre l'Agence à rembourser le surplus en raison des distorsions de concurrence que cette dotation entraînerait. C'est en effet au nom du droit européen de la concurrence que l'ordonnance met en place une organisation originale de l'activité de l'EPIC, avec l'obligation de créer des filiales consacrées à la formation des demandeurs d'emploi et des salariés. Il a en effet été estimé que seule la filialisation permettrait d'éviter que ces activités concurrentielles bénéficient en partie de la subvention pour charge de service public que l'État versera à l'EPIC. Plusieurs conditions doivent maintenant être remplies pour assurer la pérennité de ces filiales.

tandis que les formateurs resteront employés par l'EPIC. Il sera donc essentiel de définir une méthodologie de calcul incontestable des coûts que l'Agence devra facturer aux filiales pour la mise à disposition des formateurs et des locaux, faute de quoi la concurrence sur le marché de la formation sera faussée au détriment des organismes privés. Il faudra également que les filiales définissent une nouvelle offre pédagogique, adaptée aux demandes des prescripteurs, qu'il s'agisse de la région, de Pôle emploi ou des entreprises, et aux besoins des stagiaires. Elles devront résolument privilégier les outils numériques, accentuer la modularisation de leurs formations sans négliger les attentes des TPE-PME, trop rarement prises en compte aujourd'hui. Elles devront enfin adopter un pilotage de leur activité par le résultat et non par le chiffre d'affaires, comme c'était encore trop souvent le cas à l'AFPA, ce qui a pu parfois conduire dans le passé à des pratiques commerciales très contestables. Enfin, l'ordonnance règle l'imbroglio juridique relatif au patrimoine immobilier utilisé par l'AFPA qui empêchait l'assainissement de sa situation financière et obérait son développement depuis 2009, car la très grande majorité des sites de l'AFPA étaient mis à sa disposition par l'État, dans des conditions financières très avantageuses. Le Gouvernement a tout d'abord cherché, dans la loi du 24 novembre 2009, à lui transférer à titre gratuit et sans contrepartie l'intégralité de ce patrimoine. Cette disposition a été censurée l'année suivante par le Conseil constitutionnel en raison de l'absence de garanties quant au maintien de l'affectation des biens concernés à des missions de service public. La loi du 5 mars 2014 permettait quant à elle aux régions volontaires de devenir propriétaires des sites mis à la disposition de l'AFPA, sans que cette mesure rencontre néanmoins un franc succès, une seule région ayant fait ce choix. Dès lors, parmi les nombreux scénarios alternatifs élaborés, la création d'un EPIC est apparue comme la solution la plus adaptée pour tenir compte des contraintes constitutionnelles mises en lumière en 2010. De fait, le transfert des biens de l'État à une personne publique n'est pas soumis aux mêmes contraintes juridiques qu'un tel transfert à une personne privée. Ce patrimoine a toutefois été trop longtemps délaissé et mal entretenu, le propriétaire et l'occupant se renvoyant les responsabilités à ce sujet. Il convient maintenant d'évaluer précisément les besoins de rénovation et de mise aux normes et de planifier les travaux en fonction de l'activité économique de l'EPIC, ce qui n'entraînera pas des dépenses d'un montant aussi élevé que celui qui a été parfois évoqué et qui a été établi selon une méthodologie contestable. Surtout, il est maintenant impératif d'opérer la rationalisation des implantations immobilières de l'Agence, afin que celles-ci correspondent aux besoins de formation dans les territoires. L'ordonnance met également en place un mécanisme qui m'est apparu très intéressant : la mutualisation des plateaux techniques de l'EPIC au profit des acteurs du service public régional de la formation professionnelle.

ni celle du contentieux qui l'opposait à France Domaine. Les 80 millions d'euros dus aux URSSAF et au fisc, ainsi que les 140 millions d'euros réclamés au titre de l'occupation sans titre du domaine public depuis 2010 hypothèquent ses capacités de développement et seront autant d'épées de Damoclès à l'avenir. En conclusion, comme je l'ai souligné devant la commission, le changement de statut de l'AFPA constitue une condition nécessaire, mais non suffisante pour assurer la pérennité de l'activité de formation de l'Agence. La direction doit en effet mettre en place très rapidement une stratégie de développement ambitieuse. Nous faisons confiance aux autorités de tutelle, à la direction et aux salariés de l'établissement public pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire de l'AFPA. Ils ont désormais en main tous les éléments pour bâtir un outil de formation résolument tourné vers le service public et capable, à travers ses filiales, de se montrer compétitif sur le marché concurrentiel de la formation.

Avant tout, je rappelle que l'AFPA est une institution historique issue de la Libération, dont l'ambition initiale- permettre à chaque salarié, à chaque demandeur d'emploi d'accéder à une qualification diplômante partout sur le territoire national -demeure d'actualité. Ses formations de qualité, les services spécifiques qu'elle peut mobiliser au profit des publics éloignés de l'emploi, son haut niveau d'expertise et sa capacité de projection dans l'avenir devraient être reconnus et défendus par tous. Quand nous réclamons la mise en place d'une sécurité d'emploi et de formation, ce n'est pas autre chose que nous demandons aux salariés d'évoluer, de se former, de monter en qualification ou de se réorienter professionnellement. Les transformations de cette institution nous intéressent donc au premier chef,

La formation professionnelle interroge notre rapport au travail et notre modèle social ; d'ailleurs, les tensions, notamment financières, qui traversent l'AFPA, ne sont pas étrangères à ces évolutions.

Sur le fond, nous saluons les quelques avancées permises par cette ordonnance, ce qui contraste avec l'attentisme de la majorité précédente qui a failli couler l'AFPA. La crise structurelle que traverse l'AFPA ne date pas pas d'hier et 2012 aurait pu être la dernière année d'activité de la structure, il est bon de le rappeler ! Parmi ces avancées, on trouve la dévolution du patrimoine immobilier à l'AFPA, qui est désormais sécurisée juridiquement, même si de sérieuses interrogations subsistent sur les capacités financières du nouvel EPIC à en assumer l'entretien et la mise à niveau. Des aides financières ponctuelles ont permis de maintenir à flot la structure et d'éviter ainsi sa liquidation. Toutefois, la pérennité de l'AFPA est encore loin d'être assurée Son modèle économique a été bousculé par deux facteurs rappelés par le rapporteur : la décentralisation de la commande publique de formation aux régions, l'ouverture à la concurrence du champ de la formation sur le « marché de la formation. Sur ce point, mes chers collègues, nous n'oublions pas les critiques initiales de la droite, qui souhaitait en réalité libéraliser plus encore la formation professionnelle, accentuer davantage la régionalisation et la filialisation. Le projet de loi et l'ordonnance qui a été prise cet automne s'efforcent de refonder le modèle économique de l'AFPA, mais la volonté de défendre l'outil historique reste pour nous trop timide. Le Gouvernement a ainsi dû reculer face aux demandes de Bruxelles qui voyait d'un mauvais oeil les « distorsions de concurrence » qu'allait créer ce nouveau service public sur le « marché » de la formation. Résultat, on nous propose

D'ailleurs, les dotations prévues dans le projet de loi de finances pour 2017 ne prévoient de financer les missions de service public qu'à hauteur de 110 millions d'euros sur un budget de 750 millions d'euros. Plus important encore, la frontière entre activités de formation publique ou privée privée est renvoyée à une interprétation très aléatoire de la notion de « publics éloignés de l'emploi ». Le projet de loi consacre une interprétation très restrictive de cette notion, les les chômeurs de longue durée continuant à relever du marché concurrentiel, alors que leurs besoins ne sont pas fondamentalement différents de ceux des publics très éloignés de l'emploi. Ce périmètre trop étroit risque de compromettre le devenir de l'AFPA. Au final, ce seront donc les régions qui, en passant commande des formations, définiront le type de contractualisation, ce qui n'est pas pour nous rassurer En somme, le Conseil de la concurrence et le Conseil d'État ont imposé une interprétation libérale de la directive Services que le groupe CRC ne peut approuver, quand nombre de questions

au service public de l'emploi, aux côtés de Pôle emploi, et le nouveau statut d'EPIC auraient dû justifier la légalisation d'un autre mode de contractualisation entre l'AFPA et les régions ou Pôle emploi, plutôt que l'espèce de mise en concurrence abrupte qui a été retenue. À l'inverse, alors même que le plan « 500 000 formations supplémentaires », a été lancé, l'AFPA n'a bénéficié que de 18 000 entrées de stagiaires en plus en 2016, essentiellement grâce à Pôle emploi d'ailleurs, puisque les régions n'ont augmenté leurs commandes de formation que de mille places. Il est à noter que, sans ce plan, le solde net des formations financées par les régions aurait été négatif. De même, les problèmes financiers ne sont pas réglés. de la dette fiscale, sociale, des arriérés de loyers réclamés par France Domaine ? Comment l'AFPA pourra-t-elle moderniser et remettre aux normes les bâtiments que l'État lui transmet en l'état ? Ces problèmes ne sont pas résolus par cette ordonnance et pèseront sur l'avenir de la structure. Depuis deux ans, les suppressions de postes pour cause d'économies s'accélèrent, d'autres sont encore annoncées pour les années à venir. Dans ces conditions, la pérennité de la structure elle-même n'est pas complètement assurée. Voilà la vraie question ! Je sais que certains nous reprocheront d'être attachés à un modèle dépassé, mais, s'il s'agit de faire prévaloir le droit à la formation de qualité sur le droit

abstention sera un encouragement pour le Gouvernement à consulter les représentants du personnel qui ont voté de manière constante contre cette restructuration et continuent à poser des questions vitales restées malheureusement sans réponses.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous sommes réunis pour nous prononcer sur l'article unique du projet de loi qui ratifie l'ordonnance du 10 novembre 2016 portant création au sein du service public de l'emploi de l'établissement public chargé de la formation professionnelle des adultes, ordonnance prise sur le fondement de l'article 39 de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi, dite loi Rebsamen. Il s'agit donc de la transformation de l'association

Certains évoquent la décentralisation de 2004, qui confie de façon exclusive aux régions les compétences en matière de formation professionnelle, plus particulièrement le transfert des financements des formations assurées par l'AFPA, devenu effectif 2009. Cette décentralisation aurait à la fois pu être mieux accompagnée par le gouvernement de l'époque et mieux anticipée par l'AFPA. D'autres évoquent la décision du Conseil de la concurrence de 2008 qui positionne l'AFPA, comme tout opérateur de la formation professionnelle, dans le champ concurrentiel. Depuis, l'AFPA a perdu de nombreuses parts de marché, dégradant ses fondamentaux budgétaires et financiers. Ainsi, en laissant filer la situation, en laissant grossir les déficits, on peut se poser légitimement la question de la réelle volonté du gouvernement de l'époque de conserver l'AFPA. Face à cette situation insoutenable, il existait aussi- et c'est heureux ! -une autre voie. Il a donc fallu un acte politique fort de la part du nouveau gouvernement en 2012, d'abord pour inverser la spirale négative, ensuite pour créer les conditions d'une nouvelle ambition pour l'AFPA. Ce premier pas fut déterminant. Aujourd'hui, avec la ratification de cette ordonnance, nous concrétisons ce processus de refondation de l'AFPA, il est vrai au prix de certains sacrifices, qui permettent toutefois de conserver une expertise reconnue au service de la formation, de la qualification et de l'emploi. L'AFPA devient ainsi un établissement public de l'État à caractère industriel et commercial prenant le nom d'Agence pour la formation professionnelle des adultes- le sigle est

La complexité de la tâche avait sans doute été sous-estimée et l'élaboration de ce texte a buté sur des questions juridiques d'une grande complexité, au regard notamment du droit communautaire de la concurrence. Elles ont été résolues de manière satisfaisante.

l'AFPA doit analyser les besoins en compétences des bassins d'emploi, travailler à l'émergence de titres professionnels correspondant aux nouveaux métiers et assurer un appui aux opérateurs de conseil en évolution professionnelle. De manière plus spécifique, elle doit déployer des formations en développement durable et en transition énergétique. La gouvernance de l'Agence est améliorée en faisant de l'État et des régions les principaux acteurs du conseil d'administration, avec les partenaires sociaux, les représentants des salariés

RDSE votera très majoritairement ce texte. Reste que ce premier pas, aussi fondamental soit-il, n'est pas suffisant. Ce qui doit nous animer maintenant, c'est l'élaboration d'une stratégie de développement qui prenne en compte le contrat d'objectifs et de performance conclu avec l'AFPA. l'AFPA. Cela nous permettra d'aborder plus globalement la formation professionnelle dans son ensemble, qui doit s'organiser au plus près des bassins d'emploi et des entreprises, pour adapter l'offre de formation à la demande locale. La formation doit d'abord bénéficier à celles et ceux qui en ont le plus besoin, et surtout au moment où ils en ont besoin. La formation professionnelle doit aussi trouver des solutions innovantes, spécifiques pour tous ces publics. Enfin, elle doit mieux intégrer les TPE-PME ainsi que les métiers émergents. Je vois dans tout cela un puissant levier de développement piloté dans les territoires par les régions avec l'ensemble des acteurs de la formation, de l'insertion et de l'emploi. Restons confiants en l'avenir. Regardons les chiffres encourageants du second semestre 2016. L'activation du plan « 500 000 formations supplémentaires » décidé par le Gouvernement en 2016 et prolongé en 2017 porte ses fruits. C'est fondamental lorsque l'on sait que deux tiers des stagiaires retrouvent un emploi dans les six mois qui suivent leur formation. Pour conclure, je rappelle que la mise en oeuvre du compte personnel de formation, issue de la loi Travail, devrait permettre une meilleure efficience de la formation professionnelle dans les prochaines années, pour les demandeurs d'emploi comme pour les salariés, mais aussi pour tous les professionnels indépendants. Toutes ces mesures contribuent au développement de l'emploi, donc à notre développement économique. La

Prenant le relais de celles-ci, c'est en 1966 que naîtra l'Association pour la formation professionnelle des adultes. Présente sur l'ensemble du territoire, l'AFPA concentra son activité sur l'accès à la qualification des demandeurs d'emploi, puis sur la reconversion des personnes privées d'emploi. Cet opérateur parapublic était un outil de l'État dans le pilotage des politiques de formation professionnelle et de l'emploi. Ces missions étaient très largement couvertes et leur financement était principalement assuré par une subvention de l'État qui a pu atteindre 1,2 milliard d'euros en 1998. Deux événements sont venus progressivement affecter cette organisation : d'une part, la décentralisation de la formation professionnelle à l'échelle des régions en termes de commandes, d'autre part, l'ouverture du secteur de la formation professionnelle à la concurrence en application de la directive Services. Après quelques années de graves difficultés et quelques tentatives d'évolution, il s'est révélé indispensable d'engager un processus de refondation dont la transformation de l'association en EPIC peut être considérée comme une première démarche de mise en conformité. Ce changement de statut et la nette séparation entre les activités relevant de la mission de service public et celles de formation entrant dans le champ concurrentiel constituent une première étape essentielle de cette transformation. Cependant, si l'ordonnance permet de valider un nouveau cadre mieux adapté aux contraintes de l'époque, elle n'aborde pas les réformes nécessaires à la pérennisation de l'AFPA dans ses activités concurrentielles. Le changement de statut n'entraîne pas automatiquement une amélioration de la gestion. En effet, de nombreuses incertitudes demeurent sur l'organisation de l'EPIC et sur son aptitude à dégager des résultats équilibrés en termes d'exploitation.

Je m'étonne également que, avant la mise en place de ces nouvelles structures au 1 janvier 2017, le sort des dettes fiscales et sociales, lesquelles s'élèveraient à 80 millions d'euros, n'ait été réglé que par un moratoire laissant planer des incertitudes sur leur avenir.

un parc immobilier vétuste et par des charges de structure trop lourdes, comme le reconnaît la Cour des comptes, puisse connaître un redressement spectaculaire à même de garantir à lui seul la pérennité de cet outil qui capte encore environ 5 % du marché de la formation professionnelle ? Son organisation territoriale, qui a longtemps été sa force, peut être aujourd'hui un handicap si un effort d'autonomisation des structures régionales n'est pas d'une organisation déconcentrée en termes d'activités, mais centralisée en termes de moyens, de ressources et de pouvoir de décision, ne favorise pas la responsabilisation, la réactivité ni l'adaptation rapide aux besoins de marchés qui sont souvent devenus régionaux. ! L'emploi du terme « marché » peut paraître choquant pour un outil parapublic, mais il correspond aujourd'hui à une réalité puisque, par exemple, les régions sont tenues de procéder par appels d'offres pour choisir leurs prestataires. L'AFPA est-elle aujourd'hui en mesure d'affronter la concurrence du secteur privé ? La question reste posée et c'est l'avenir qui nous donnera la réponse.

Reconnaissant le caractère indispensable de la transformation de l'association en EPIC, mais mesurant la très grande fragilité de cette évolution en raison des incertitudes et des inquiétudes évoquées précédemment, le groupe de l'UDI-UC ne s'opposera pas à la ratification de cette ordonnance. La parole

Comme cela a été rappelé, le Gouvernement avait été habilité à prendre cette ordonnance par la loi Rebsamen du 17 août 2015. Comme notre rapporteur, je fais le constat que le Gouvernement a respecté l'objet et les délais fixés par l'habilitation.

définir les conditions de dévolution d'actifs immobiliers de l'État à l'EPIC et de préciser les conditions du transfert des biens, droits et obligations de l'association à cet établissement. Ainsi, l'association a été dissoute le 22 décembre dernier et l'EPIC a vu le jour le 1 janvier 2017. Cet établissement se nomme désormais Agence pour la formation professionnelle des adultes, ce qui a permis de préserver le sigle AFPA. Sa mission de service public a été précisée et deux filiales ont été créées pour accueillir les activités de formation professionnelle des demandeurs d'emploi soumises au droit européen de la concurrence. Par ailleurs, 116 sites d'une valeur estimée à 410 millions d'euros ont été transférés gratuitement à l'EPIC. Le Gouvernement nous dit avoir tout mis en oeuvre, tant financièrement que juridiquement, pour sauvegarder et renforcer l'AFPA.

Les efforts du Gouvernement ont permis, pour l'instant, de sauvegarder un opérateur public de formation professionnelle.

le patrimoine alloué à l'Agence nécessite d'importants travaux de désamiantage, de rénovation thermique et de mise aux normes en Si le Gouvernement conteste le chiffre de 1,2 milliard d'euros avancé par la direction de l'AFPA et par les syndicats, il ne fait aucun doute que les travaux devant être engagés coûteront des dizaines, voire des centaines de millions d'euros. parle pas du contentieux locatif, pour lequel France Domaine réclame 130 millions d'euros à l'AFPA. la réforme ne permet en rien de résorber le déficit budgétaire structurel de l'association, dont le chiffre d'affaires ne fait que décroître, ce qui entraîne la suppression de personnels et donc un déficit d'activité, lequel fait baisser le chiffre d'affaires, sans que l'on voie comment enrayer ce cercle vicieux. Enfin, les règles européennes en matière de concurrence et l'ambiguïté de la définition du service public de l'emploi dans le texte même de l'ordonnance interdisent à l'État de financer l'Agence au-delà des 110 millions qu'il lui verse annuellement, ce montant étant sans doute appelé à diminuer. Au passage, le groupe écologiste regrette profondément que les actions de formation en matière de développement durable et de transition énergétique ne soient pas considérées comme relevant d'une mission de service public et qu'elles ne fassent donc pas l'objet d'une dotation de l'État. Cela nous semble contradictoire avec l'article 2 de la loi relative à la transition énergétique Face à ce triple constat, le doute s'installe. Comment, dans ces conditions, préserver le service public de la formation professionnelle ?

lancer sans attendre l'appel d'offres national sur les formations rares et émergentes rendu possible par la loi Sapin II, harmoniser les appels d'offres de formation professionnelle d'une région à l'autre afin de diminuer le volume de tâches administratives de l'Agence et de ses concurrents du envisager d'accorder à l'AFPA une délégation de service public pour pérenniser un certain nombre d'activités, sans entraver le droit à la concurrence. Il reviendra également à l'Agence de rationaliser son nouveau patrimoine immobilier,

dit, une incertitude planait sur le patrimoine immobilier de l'AFPA après la censure du Conseil constitutionnel. Enfin, pour ne rien arranger- et j'arrêterai là ce sombre tableau -, le transfert des personnels chargés de l'orientation des demandeurs d'emploi

ont apporté un bol d'air à l'AFPA, mais il fallait lui donner une nouvelle assise juridique, clarifier ses missions, lesquelles doivent être en phase avec les mutations en cours dans notre économie. Tel est l'objet de l'ordonnance.

1,1 million d'actions de formation, dont 300 000 pour les publics prioritaires. Ce plan a permis une très nette accélération de l'activité de l'AFPA à partir du mois de septembre 2016

L'ordonnance clarifie la situation juridique, les missions et la gouvernance de l'Agence. Elle règle le transfert du parc immobilier. Cela suffira-t-il à répondre à une situation critique ? Bien sûr que non. L'AFPA devra augmenter son activité,

L'avenir de l'AFPA est également conditionné à celui de la formation professionnelle. Les choix qui seront faits lors du printemps électoral seront déterminants.

Le nombre de comptes ouverts a augmenté de 53 % : 12,3 millions d'heures ont été mobilisées. La loi relative a permis de doubler, à partir du 1 janvier 2017, les droits à la formation inscrits dans le compte personnel d'activité des personnes peu qualifiées et a institué un mécanisme d'abondement des droits à la formation pour les jeunes sans qualification. Ces efforts doivent s'intensifier, notamment en direction des publics prioritaires, au premier rang desquels figurent les chômeurs, car le système actuel,

n'est pas un révolutionnaire, s'exprimait ainsi sur la bonne utilisation des 30 milliards d'euros consacrés à la formation professionnelle : « Il y aurait beaucoup à faire pour rendre leur emploi efficace. » Il ajoutait : « La gouvernance n'est pas assurée, il y a plusieurs pilotes dans l'avion. »

un accès universel à la formation avec accompagnement personnalisé, assorti pour le bénéficiaire d'une obligation d'assiduité vérifiable- lisez la synthèse du rapport de la Cour - ; un accès diversifié allant des formations courtes, permettant de maîtriser une technique indispensable, à des formations longues en vue d'une reconversion professionnelle ;

une faute politique très lourde

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, ce projet de loi s'inscrit dans le prolongement de plusieurs réformes engagées par la majorité précédente, dans une logique de décentralisation et de rationalisation de la formation professionnelle. Ainsi, en 2004, l'État transférait aux régions une compétence générale en matière de formation professionnelle, ce qui impacta le fonctionnement de l'AFPA, désormais soumise au droit de la concurrence et aux exigences des conseils régionaux, des appels d'offres. Ce nouveau cadre allait provoquer un enchaînement d'aménagements juridiques, dont j'ai pu constater la complexité. S'est tout d'abord posée la question du partage des missions de l'AFPA.

Il devenait en effet nécessaire de rationaliser les services et donc de regrouper au sein de Pôle emploi les fonctions d'orientation proposées aux demandeurs d'emploi afin de leur éviter le parcours du combattant que représente la dispersion des structures administratives. J'en profite pour rappeler que, à l'origine, Pôle emploi a été créé pour faciliter le parcours des chômeurs et des personnes à la recherche d'un emploi. Le transfert des personnels d'orientation de l'AFPA répondait également à un impératif juridique, car le Conseil de la concurrence craignait une atteinte à la concurrence si l'AFPA orientait les demandeurs d'emploi vers ses propres centres de formation.

notre rapporteur, l'État a en effet souhaité transférer à titre gratuit à l'AFPA les biens immobiliers qu'elle louait, soit 158 centres de formation, afin de la doter des moyens de son autonomie et de lui permettre de faire face à ses mutations. professionnelle, cette dévolution s'est heurtée à la censure du Conseil constitutionnel, qui a considéré qu'il s'agissait de biens publics protégés et que rien ne garantissait que ces biens demeurent affectés au service public. droit communautaire, l'opération risquait également d'apparaître comme une aide d'État. En 2014, le Gouvernement a cherché à tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel en mettant en place un mécanisme de transfert à titre gratuit aux régions,

Ces incertitudes ont eu des conséquences défavorables sur la gestion de l'AFPA, l'exposant notamment à devoir verser des arriérés de paiement sur ses redevances. Il était donc plus que temps de proposer une solution satisfaisante au regard du droit constitutionnel et du droit communautaire. J'ai aussi été rapporteur de la loi relative au dialogue social qui comportait l'habilitation à légiférer par la présente ordonnance afin de transformer l'AFPA en un établissement public à caractère industriel et commercial doté d'une mission de service public.

en mettant en place la décentralisation de la formation professionnelle et en soumettant l'AFPA à un régime concurrentiel, était à l'origine de ses difficultés financières, ou tout au moins qu'elle ne les avait pas anticipées.

prévue pour le 1 janvier 2009 pour le transfert progressif aux régions de l'organisation et du financement des stages de l'AFPA », mais que « le système de subvention prolongée conclu avec les régions n'avait pas été mis à profit pour engager une réforme progressive du financement des stages de l'AFPA avant sa confrontation à une mise en concurrence effective ». Pour expliquer ces difficultés strictement internes à l'AFPA, la Cour a évoqué

professionnelles finançant par ailleurs leurs propres systèmes de formation -, ainsi que « des conflits récurrents avec les représentants syndicaux sur les plans sociaux successifs, puis entre le président de l'association et le directeur général général ». Outre ces problèmes de gouvernance, l'AFPA a tardé à intégrer le rôle de la région dans la formation professionnelle, et son organisation territoriale n'a pas évolué, alors que la nouvelle logique de marché public reposait non non sur une stratégie unique pour l'ensemble du territoire, mais sur des modalités propres à chaque région. Une absence systématique d'analyse du marché l'a également empêchée de gérer ses problèmes de transition d'une structure subventionnée par l'État à un organisme essentiellement commercial. La Cour des comptes a également souligné une diminution trop lente des effectifs, une politique de gestion des ressources humaines insuffisamment rigoureuse, un manque de mobilité des personnels, des problèmes de facturation, ainsi que la réduction tardive des charges de fonctionnement, contribuant à dégrader les comptes de l'AFPA. Je tenais à rappeler ces faits qui, vous le constatez, ont peu à voir avec une supposée inaction de l'État. Toujours est-il que l'AFPA dispose, selon moi, d'atouts importants, en particulier pour faciliter un retour durable des demandeurs d'emploi sur le marché du travail- ce qui est l'objectif principal -, grâce à son outil de formation à son savoir-faire dans le domaine de l'accompagnement des stagiaires. Il ne faut pas oublier que la moitié des stagiaires demandeurs d'emploi ayant obtenu un titre professionnel sont en situation d'emploi six mois après la fin de leur formation. Aujourd'hui, en rendant l'AFPA maître de ses principaux outils et en lui octroyant un statut plus conforme au cadre concurrentiel, nous espérons la replacer sur une trajectoire viable et préserver ses compétences et son savoir-faire. Le groupe Les Républicains joindra donc ces voix à celle du rapporteur et à celles de la plupart des groupes en faveur d'une adoption conforme du présent texte, souhaitant sa mise en oeuvre rapide. Pour ma part, j'espère que ce sera la dernière fois qu'une loi sera nécessaire pour régler les problèmes de l'AFPA.

M. le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de réunion d'une commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité publique. En conséquence, les nominations intervenues lors de En conséquence, les nominations intervenues lors de notre séance du mercredi 8 février prennent effet.

et le soir : Conclusions des commissions mixtes paritaires sur le projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2016-966 du 15 juillet 2016 portant simplification des procédures mises en oeuvre par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé